Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des lois a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement suivie d'un débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution. Mes chers collègues,

Monsieur le Premier ministre, vous avez reçu Monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire l'immense honneur et la grande émotion que je ressens au moment de m'exprimer devant la Haute Assemblée que vous formez. Si j'ai tenu à présenter la politique de mon gouvernement devant le Sénat, c'est avant tout pour marquer mon attachement

Devant vous, comme hier devant l'Assemblée nationale, je veux témoigner de notre profond attachement à notre système représentatif.

la gravité du contexte national, européen et international dans lequel j'ai accédé à cette haute responsabilité. Je mesure que je dirige un gouvernement de crise, donc un gouvernement de combat.

Je tiens à préciser au Sénat les intentions du Gouvernement dans la période actuelle, marquée- vous le savez -à la fois par une forte activité de l'épidémie dans certaines parties du monde

ne visent pas tant à répondre, ici, en métropole, à une situation d'urgence, qu'à nous inscrire dans une logique préventive.

Mais nous devons être pragmatiques : sans certitude absolue qu'une telle action soit possible, j'ai décidé que nous allions amplifier les mesures de contrôle sanitaire à l'arrivée sur le territoire national, dans les ports et les aéroports.

et le point le plus positif, c'est que leur résultat, quand ils sont pratiqués, demeure très largement favorable. En tout cas, de tests positifs est très nettement inférieur aux modélisations réalisées au mois de mai dernier, ce qui témoigne sans doute de l'efficacité de la politique conduite.

pour les réaliser, notamment depuis que les techniciens de laboratoire ont été autorisés à effectuer les prélèvements ; mais nos concitoyens ne se font pas suffisamment tester, sont sensibles à l'ambiance générale- on affirme que l'épidémie est maîtrisée, ce qui est le cas. Il faut donc lever tous les obstacles, y compris psychologiques, qui expliquent cette situation. le Président de la République a annoncé la fin des prescriptions médicales obligatoires pour se faire tester. En outre, j'ai demandé que nous accélérions

enfin, le port du masque constitue, avec le respect des gestes dits « barrières », une mesure de prévention et de protection efficace. J'ai donc proposé que l'obligation de le porter soit renforcée dans tous les établissements recevant du public clos, en particulier- ce n'est pas le cas aujourd'hui -les commerces. Cette mesure nécessite un décret, alors que, dans les locaux dits « professionnels », elle suppose une évolution des protocoles sanitaires régissant les activités concernées. Nous envisagions une entrée en vigueur de ces dispositions le 1 août

paraissait tardive ou suscitait quelques interrogations : le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine. j'ai demandé aux ministres chargés de la santé, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de donner très rapidement des indications précises aux familles et au corps enseignant

heure. Vous le savez, chargé par le précédent gouvernement de préparer le déconfinement, j'avais recommandé que le couple maire-préfet de département soit placé au coeur du dispositif, ce qui fut fait. J'avais également suggéré que l'on soutienne les collectivités territoriales dans leur politique d'acquisition de masques pour conforter et démultiplier nos actions, ce qui fut fait également.

nos finances publiques et nos finances sociales, venant fragiliser notre modèle. Elle nous rappelle également l'ampleur du défi écologique. les sénateurs, il est des heures où l'ensemble des forces vives d'un pays doivent plus que jamais se rassembler. Ma conviction est que nous sommes précisément dans un tel moment. l'esprit de dialogue, la volonté de dépasser les postures et les clivages ; et ce sont, je le sais, des principes qui vous sont chers. À ce titre, les Français eux-mêmes nous ont donné l'exemple. Ils ont été solidaires et résilients face à la crise sanitaire. Nous devons prendre collectivement la mesure de la situation. Si nous ne réagissons pas, elle pourrait accentuer les fractures qui traversent notre pays et menacer notre unité, déjà bien mise à mal, notamment en aggravant les fractures territoriales. crise à bras-le-corps, protéger les Français, reconstruire notre économie et, au-delà, conforter notre pacte républicain tels sont les défis qui se présentent devant moi et devant le gouvernement que je conduis. Mon discours de politique générale, hier devant l'Assemblée nationale, a été lu devant vous par M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Je ne reviendrai donc pas en détail sur l'ensemble des mesures que j'ai évoquées. Merci ! Vous l'avez compris : ma conviction est que, pour réussir, nous devons changer nos façons de faire. Il faut le dire et le réaffirmer : l'État a un rôle majeur, mais il ne pourra agir seul. Il devra fédérer les bonnes volontés, mobiliser toutes les énergies et faire confiance à tous ses partenaires, à commencer par les collectivités, que vous représentez.

l'exercice de la responsabilité politique ne peut s'arrêter aux intentions, si louables et ambitieuses soient-elles. Rien ne vaut sans l'obsession du résultat et de l'impact sur la vie de nos concitoyens. J'ai rappelé hier cette phrase célèbre : « L'intendance suivra. » l'intendance ne suit pas, en tout cas pas toujours, et même de moins en moins, alors même que cela devrait être la priorité. La mise en oeuvre, l'exécution, les conditions de réalisation doivent entrer clairement dans le champ de la politique et ne plus être considérées comme de simples sujets triviaux et techniques. Je vous le concède volontiers : il s'agit là d'un choc culturel dans un pays où, depuis le siècle des Lumières, le débat d'idées, l'invocation des grands principes et le maniement des concepts monopolisent

C'est surtout par l'exécution, par la charge de la preuve, que se reconstruira la confiance, dont les responsables publics ont tant besoin et qui, vous le savez comme moi, s'est fortement altérée. Pour réussir, nous ne pouvons donc pas nous contenter de fixer un cadre juridique national. Nous devons nous impliquer dans le déploiement, dans la mise en oeuvre des politiques publiques au sein des territoires, pour les adapter à la vie des gens dans nos régions, nos départements, nos cantons, nos communes et nos quartiers.

La République territoriale, c'est l'unité dans la diversité. Je compte sur vous, durant les 600 jours qu'il nous reste, pour m'aider dans un esprit de concorde, parce que, si la défiance progresse encore, elle nous emportera tous. Mesdames, messieurs les sénateurs, la bataille de l'emploi sera la priorité Pour 2020, nous prévoyons à ce jour une récession de 11 %, soit la récession la plus sévère depuis que les comptes nationaux ont été créés. Derrière les données comptables, il y a des drames humains, des territoires meurtris. Tout cela, nous devons le prévoir, l'accompagner, le soulager, et nous devons aller plus loin. Nous devons nous saisir de cette situation pour reconvertir notre économie, nos travailleurs et nos salariés ; pour les rendre plus forts et plus compétitifs ; pour les orienter davantage vers une croissance durable et respectueuse de l'environnement. Tel est l'objectif

Vous en connaissez les vecteurs : le chômage partiel, les prêts garantis par l'État et le fonds de solidarité, qui ont représenté un effort global et massif de près de 500 milliards d'euros.

; ses résultats ont été salués par tous, à commencer par le peuple français. Très vite et très tôt, nous avons également mis en place des plans sectoriels très ambitieux dans le tourisme, l'aéronautique, l'automobile, la culture, le commerce, le bâtiment et les

semblent indiquer une reprise plus rapide que prévu. Mais grâce à qui ? En particulier, la consommation des ménages affiche une reprise solide depuis la fin du confinement.

protéger les Français, reconstruire et moderniser la France. En particulier, en prolongeant les dispositifs d'activité partielle, nous mettons tout en oeuvre pour préserver l'emploi et les salaires dans les entreprises les plus touchées par la crise.

Il n'est pas question de laisser s'installer l'idée d'une génération sacrifiée à cause de cette crise. Pour cela, nous allons engager des mesures fortes.

très fortement le coût du travail pour faciliter l'embauche des jeunes. Parallèlement, nous allons développer massivement, dans des proportions qui n'ont jamais été atteintes, les dispositifs d'insertion, en particulier à l'intention des jeunes les plus en difficulté. Le service civique, au service de l'engagement des jeunes et de leur insertion, sera considérablement renforcé. Ce sera aussi l'une des manières de soutenir nos associations et leurs vingt millions de bénévoles, qui- personne ne l'oublie -sont un atout majeur pour renforcer la cohésion nationale et le lien social dans notre pays. À l'université, la crise a agi comme révélateur des difficultés que rencontrent encore de trop nombreux étudiants. Nous avons décidé de geler les droits d'inscription et de porter à 1 euro le prix des repas dans les restaurants universitaires pour les étudiants boursiers.

ce dernier exige, de notre part, des interventions fortes et nouvelles : il faut améliorer son fonctionnement et mieux en garantir les équilibres dans la durée.

dans un contexte de tension extrême, qui- nous devons bien le reconnaître -préexistait à la crise du covid.

Au-delà de ces moyens financiers, il faut améliorer le fonctionnement quotidien des structures en leur donnant davantage de souplesse : elles doivent pouvoir déroger à certains cadres nationaux sur des questions de gouvernance interne, d'organisation et de modalités de temps de travail. favoriser davantage les logiques de décloisonnement entre ville et hôpital, à l'échelle des territoires. Enfin, il faut permettre aux collectivités d'être davantage parties prenantes des stratégies d'investissement et d'organisation des soins, au niveau tant des agences régionales de santé que des établissements eux-mêmes. À

conclus avec l'État et les structures de soins, et avec à la clé, je le répète, une participation accrue des élus à la gouvernance du système. Je n'ignore pas que l'autre question majeure que nous posent nos concitoyens dans le domaine de la santé a trait à la difficulté qu'ils rencontrent pour accéder à un médecin, généraliste ou spécialiste, notamment en ville.

Nous devons agir de manière pragmatique, pour être efficaces à court terme. La seule solution, en tout cas l'une des principales, consiste à permettre aux médecins en exercice de travailler dans de meilleures conditions, au sein d'organisations plus collectives, en favorisant la délégation de plus de tâches, en les dotant d'assistants médicaux et en les allégeant des trop nombreuses charges administratives, qui leur prennent du temps. L'autre priorité est de recourir davantage à la télémédecine, dont j'ai pu constater dans mon territoire

ampleur. Il nous appartient maintenant de consolider et de sécuriser sa place parmi les pratiques médicales. Nous ne retrouverons pas l'unité sans une attention accrue aux plus vulnérables d'entre nous. Davantage touchés par la crise sanitaire, ils seront également, avec les jeunes, les plus fortement affectés par la crise économique, à commencer par les personnes en situation de handicap. Nous réunirons une Conférence nationale du handicap consacrée à ces sujets. Mesdames, messieurs les sénateurs, consolider notre modèle de protection sociale, c'est aussi prendre les mesures nécessaires pour assurer sa pérennité. En matière de retraites, la crise nous invite plus que jamais à poursuivre nos objectifs vers un système plus juste et plus équitable, notamment pour les femmes et les travailleurs modestes. Ce système passe par la création d'un régime universel,

Dans le même temps, je pense que nous devons entendre les inquiétudes et les incompréhensions exprimées par nos concitoyens s'agissant de certaines modalités du projet dont le Parlement a été saisi. Je proposerai donc aux partenaires sociaux, comme aux parlementaires, que, sur les bases que je viens d'indiquer, la concertation reprenne rapidement, afin d'améliorer le contenu et la lisibilité de cette réforme nécessaire, en la distinguant très clairement de tout enjeu d'ajustement paramétrique- pour employer une formule technocratique -des régimes existants. En effet, je suis convaincu que, s'agissant d'une réforme qui nous engagera pour des décennies,

de la première phase de réforme des régimes spéciaux, décidée en 2007. Au-delà de la retraite,

doit aboutir à un projet de loi, dont vous serez saisis au premier semestre de l'année prochaine. je demanderai demain aux partenaires sociaux de se saisir, avec l'État, des questions liées à l'équilibre de l'ensemble des régimes de protection sociale, profondément affectés par la crise. L'unité suppose aussi que l'État demeure le garant de l'ordre républicain. L'État doit être le même pour tous : nous ne tolérerons aucune zone de non-droit À tous nos concitoyens, je veux affirmer notre totale détermination à assurer leur sécurité. Je le disais hier à l'Assemblée nationale et je le répète devant vous ce matin : nous ne montrerons aucune faiblesse contre tous ceux qui s'en prennent à l'ordre public, tentent de fracturer le pays entre communautés et portent atteinte aux valeurs cardinales de la laïcité. À nos policiers et gendarmes j'exprime, au nom de la Nation, mon profond respect et ma gratitude. Incarnant l'ordre républicain, ils exercent leur mission dans des conditions parfois extrêmement délicates. Je veillerai, avec M. le ministre de l'intérieur, à ce qu'ils obtiennent les moyens matériels et humains nécessaires pour conduire leurs missions et à ce qu'ils puissent être présents là où ils sont attendus, sur le terrain, en étant déchargés au maximum de tâches administratives qu'on le dit ... Je ne puis parler de ceux qui protègent les Français sans évoquer le rôle fondamental de nos armées.

qu'un effort exceptionnel de la Nation a été décidé pour renforcer leur efficacité.

que les forces de police et de gendarmerie reçoivent la reconnaissance et les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission, mais il faut aussi, et peut-être surtout,

Il en résulte que l'action des forces de l'ordre reste parfois sans suite et que des situations d'impunité sont ressenties comme particulièrement inacceptables par nos concitoyens et les élus de territoire- les maires au premier chef. Vous avez voté une loi de programmation et de réforme de la justice ; j'entends en accélérer la mise en oeuvre, en réorientant par redéploiement, dès des moyens affectés au budget de ce ministère, notamment pour rendre plus rapide et effective la réponse judiciaire, améliorer la politique des peines, garantir la dignité et la réinsertion des prisonniers et moderniser le fonctionnement des juridictions.

Il faut donc aller au coeur du dispositif : c'est le devoir de l'État, c'est l'intention de mon gouvernement ! Chiche ! Renforcer la confiance,

des sceaux est particulièrement attaché. Aucune forme de violence ne peut être tolérée ! La lutte contre les violences conjugales sera l'une des grandes priorités de la politique pénale du Gouvernement. Faire régner l'ordre, rendre la justice : ce sont les valeurs cardinales de l'État. Mesdames, messieurs les sénateurs, parlant du pacte républicain et de l'unité de la Nation, je tiens à marquer mon attachement profond à l'école de la République. Fils d'institutrice, je sais ce que je dois à la méritocratie républicaine. Je veux d'ailleurs dire toute mon admiration au corps enseignant. Depuis trois ans, une profonde refondation de l'école a été engagée ; nous la poursuivrons, en tirant, là aussi, les enseignements de la crise et en concentrant notre action sur les enfants qui ont décroché durant le confinement. Ainsi, dès le début de l'année scolaire, les professeurs veilleront à identifier les besoins de chaque élève, grâce à des évaluations nationales. Chaque famille qui en fera la demande pourra bénéficier pour son enfant d'un programme personnalisé de soutien scolaire au cours du

que mon gouvernement s'appuiera sur les territoires pour conduire sa politique. C'est une question de respect ; c'est surtout une question d'efficacité. l'État, je le répète, est le garant des fonctions régaliennes qui scellent l'unité de la Nation, pour l'ensemble des grandes transitions écologiques, économiques et sociales, ce sont les acteurs territoriaux qui doivent être à la manoeuvre L'État et les collectivités territoriales ont la République en partage : ils sont les partenaires indispensables de la réussite de nos politiques publiques. Dès les premiers jours qui ont suivi ma prise de fonction, j'ai rencontré l'ensemble des associations représentatives des collectivités

Toutes les collectivités territoriales y auront une part essentielle. Nous devons rapidement achever de régler avec elles les questions liées aux conséquences de la crise sur leurs finances,

puissent, parce que c'est dans leurs gènes, investir, former et agir de la manière la plus massive possible, mais en cohérence avec nous.

Le plan de relance prévoit d'ailleurs de soutenir les interventions des collectivités territoriales dans leur champ de compétences. impérativement redonner du sens et surtout de la chair au futur contrat de plan et de territoire. Je voudrais insister devant vous sur deux chantiers majeurs, qui illustreront cet engagement partagé.

1,5 milliard d'euros supplémentaires. Nous nous fixons l'objectif de 200 000 places supplémentaires pouvant être ouvertes en 2021 au bénéfice des jeunes et des demandeurs d'emploi. Qui peut imaginer que nous pourrions construire ce plan sans le concours des régions, compétentes au premier chef en la matière ? Bravo ! Très bien ! Nous devons également poursuivre l'effort de reconquête industrielle, au travers du programme « Territoires d'industrie », largement décliné par les régions. autre priorité essentielle est la transition écologique. Cette dernière réussira d'autant mieux qu'elle reposera sur une mise en oeuvre partagée et territorialisée.

tout d'abord, dans le bâtiment et les transports. Nous investirons aussi dans les technologies vertes de demain, comme l'hydrogène, mais aussi pour mieux recycler et moins gaspiller. Accélérer la transition écologique, c'est investir également en faveur d'une offre d'alimentation saine et durable, pour que tous les Français, même les plus fragiles, aient accès à une alimentation de qualité. nous allons aussi protéger les terres agricoles. À cet égard, j'ai annoncé hier, à l'Assemblée nationale, notre volonté de décréter un moratoire pour tout projet nouveau d'installation de centres commerciaux dans les zones périurbaines. Nous définirons, en concertation avec vous et toutes les parties prenantes, de nouvelles règles d'autorisation d'exploitation commerciale. Surtout, pour réussir cette reconstruction, nous allons donner davantage de liberté aux territoires et aux collectivités

ne peuvent douter que ces propositions feront l'objet de ma part d'un examen très attentif et très bienveillant.

Jacqueline Gourault, reprend les nombreuses concertations lancées en janvier dernier, dans le cadre de la préparation du futur projet de loi dit « 3D », pour décentralisation, déconcentration, différenciation.

aboutira à une prochaine Conférence nationale des territoires, où nous annoncerons clairement nos intentions. Tout d'abord, nous allons consacrer le droit à la différenciation dans une loi organique. Concrètement, développer la différenciation, c'est avant tout faciliter l'expérimentation. Oui, des réponses différentes doivent être apportées à des situations différentes dans notre pays, construit depuis plus de deux siècles sur l'uniformisation, c'est une révolution ! Dès la fin de ce mois, un projet de loi organique sera présenté en conseil des ministres, qui donnera un nouveau cadre aux expérimentations menées par les collectivités territoriales pour qu'elles ouvrent la voie à une différenciation durable. Un autre projet de loi viendra consacrer et donner de l'effectivité à ces trois principes : différenciation, décentralisation, déconcentration. Donner plus de liberté aux collectivités territoriales, c'est aussi faire évoluer profondément l'organisation interne de l'État. est nécessaire aussi pour rendre l'État plus proche des concitoyens. Je le dis pour l'avoir vécu : l'État s'est trop éloigné.

Nous rendrons rapidement plus cohérente et plus efficace l'organisation de l'État, en particulier au niveau du département. Les moyens de l'État seront confortés pour l'action quotidienne, dès le projet de loi de finances pour 2021.

C'est une révolution dont je vous prie de mesurer qu'elle va me causer beaucoup de soucis

-pour pérenniser les dispositifs de dérogation et de simplification administrative adoptés par ordonnances à la faveur de la crise sanitaire.

ampleur, justifiera que nous allions encore plus loin, encore plus fort, dans les démarches de simplification, qu'il s'agisse du droit de la commande publique, des autorisations

une mine de propositions en la matière. Mesdames, messieurs les sénateurs,

Je souhaite vous faire partager ma conviction que la priorité des priorités, c'est de trouver ou retrouver le chemin d'un développement économique du monde rural. En réalité, si les services publics y ont fermé au cours des dernières années, c'est parce que la population y a diminué. Et si la population y a diminué, c'est d'abord parce que l'économie et l'emploi dans notre pays se concentrent désormais dans les très grandes agglomérations.

Doit-on conserver des routes nationales, que l'État a bien du mal à entretenir et qu'il ne développe plus ?

dans leur rôle de responsables de toutes les mobilités, en envisageant des routes structurantes d'intérêt régional ? On refile

Il s'agit de faire de toutes nos villes, petites et moyennes, des lieux plus attractifs, exemplaires, dotés de services essentiels et où il fait bon vivre. De même, j'ai fixé à mon gouvernement des objectifs précis et quantifiés s'agissant du plan de rénovation urbaine et des 450 quartiers de la politique de la ville.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la République ne serait rien sans les territoires qui la composent, dans leur diversité et leur insondable richesse. Cette diversité, croyez-moi, je la connais bien Fils du Gers- un territoire rural -, élu dans les Pyrénées orientales- un territoire éloigné je suis surtout un enfant de la République, que je m'efforce de servir avec passion. Je suis persuadé que cette diversité de la France, qu'exprimait avec admiration Fernand Braudel au soir de sa vie, est plus que jamais un chemin d'espérance. C'est en tout cas le sens de l'action que j'entends mener à la tête du Gouvernement que j'ai l'honneur de diriger, sous l'autorité du Président de la République. C'est le sens de l'engagement qui est le mien depuis de nombreuses années, engagement porté dans les différentes responsabilités publiques et mandats démocratiques que j'ai exercés au service de nos concitoyens. C'est surtout le sens de la mobilisation collective qui doit être la nôtre dans les circonstances, très difficiles, traversées C'est le sens de l'invitation que j'adresse à toutes les forces démocratiques, à toutes les forces vives, à tous les territoires.

l'argent a coulé à flots ; pourtant, notre économie et l'emploi risquent d'être au coeur d'une situation explosive. N'ayant que cinq minutes de temps de parole, monsieur le Premier ministre, je ne vais pas aborder tous les sujets. d'abord, je souhaite que vous sachiez trouver les bonnes solutions pour que le secteur de la santé soit traité avec efficacité et humanité. Tout n'est pas affaire d'argent, mais notre pays est confronté à un double enjeu être prêt à affronter un retour de la pandémie et ne pas laisser de côté, pour ce motif, ceux qui ont un droit légitime à être soignés, quel que soit le besoin. Rapporteur du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, j'ai rédigé de nombreux rapports sur la valorisation de la recherche. J'espère que Mme la ministre Frédérique Vidal saura trouver auprès de vous les moyens d'une loi dynamique, dont nous attendons beaucoup. L'avenir de la France dépend, en effet, de notre capacité à mobiliser les énergies créatrices et, surtout, transformer en réalité économique le formidable réservoir de notre excellence scientifique.

Je pense pouvoir faire quelques observations, n'ayant d'autre valeur que d'être le fruit d'une modeste expérience ... Des discours, des bonnes intentions et des analyses pertinentes, j'en ai entendus beaucoup Rien ne vaut la réalité des faits ; c'est par les actes que l'on juge une politique. La politique, c'est comme l'art de la guerre : tout dépend de l'exécution. Une bonne exécution est tout d'abord cohérente. La cohérence suppose que l'on se concentre sur l'essentiel : la priorité des priorités, c'est l'économie, l'emploi, l'avenir des jeunes. Vous avez proposé des mesures qui vont dans le bon sens. Seront-elles assez rapidement opérationnelles ? Prenons l'exemple des jeunes censés intégrer le marché de l'emploi. Vous avancez des mesures visant à alléger les charges des entreprises. Mais celles-ci n'ont plus de trésorerie Ce n'est pas à la hauteur de l'enjeu. Cela ne provoquera pas le déclic immédiat et enthousiasmant qui serait nécessaire. Il faudrait plutôt que chaque entreprise puisse embaucher un ou plusieurs jeunes, à proportion de son effectif, avec un financement de l'État pendant un an.

aux entreprises ayant des carnets de commandes- cela ne vous coûtera rien. Mettez-les en situation de s'adapter à une demande multiforme. Libérez les heures supplémentaires- il n'est pas nécessaire de les défiscaliser ! L'avenir de notre pays dépendra de ce que vous serez capable de faire à la rentrée, comme nos voisins européens. Ne polluez pas ce combat par des décisions qui ne peuvent que nous diviser et, donc, diminuer notre effort ! Nous ne souhaitons pas votre échec, monsieur le Premier ministre. Il vous revient la responsabilité de savoir écouter, même les anciens qui tirent leur révérence

s'opposer à la loi du marché qui domine tous les secteurs de la vie, y compris la santé ; faire sauter les verrous budgétaires libéraux qui, jusqu'à la dernière loi de finances et à la présentation du projet de loi sur les retraites, étaient les marqueurs du discours présidentiel. La crise sanitaire, violente, a cruellement mis en évidence le grand désordre suscité par la mondialisation financière. Le capitalisme, dans une fuite en avant cupide et inhumaine, a porté une lourde part de responsabilité dans les difficultés de notre pays à faire face à l'épidémie. Nos concitoyens ont découvert avec stupeur la délocalisation massive de la production de médicaments, de masques et de réanimateurs. Voilà pourtant des années certains, dont nous étions, soulignaient les ravages des délocalisations, cette absurdité sociale au service du profit des actionnaires. Leur terrible Leur terrible impact, appliqué au système de santé, a convaincu une grande majorité de nos concitoyens qu'il fallait changer de logiciel pour notre économie et, sans doute, pour notre société. Monsieur le Premier ministre, ni le Président de la République, qui voulait se réinventer, ni vous-même ne nous avez convaincus de votre volonté de rompre avec un système, dans lequel l'argent roi prévaut sur l'humain. La crise économique est là ; elle aussi est violente. Bien sûr, vous mettez l'orthodoxie budgétaire dictée par les règles européennes entre parenthèses, car vous avez besoin de sommes considérables pour faire face au choc actuel. Néanmoins, sur le fond, vous gardez ensemble le cap. Et ce cap, c'est l'adaptation de notre pays à la mondialisation financière fondant le système auquel vous adhérez- en dépit, monsieur le Premier ministre, de vos références à un gaullisme social désuet. désuétude, car la puissance publique a été dévorée par le marché, année après année, privatisation après privatisation ! J'ai cette impression fugace, mais bien détestable

M. Macron, dans un exercice de repentance bien appuyé, reconnaissait s'être trompé, avoir porté des mesures injustes. Mais, en même temps, il vantait les mérites de sa politique, dus, selon lui, au projet qui a justement dressé le peuple contre lui. Réforme de la SNCF, réforme du travail, politique fiscale : voilà les bons points qu'il s'est distribués le 14 juillet dernier. Le cap, c'est le libéralisme sans frein. La réforme des retraites est, à ce titre, symbolique. Vous l'exhumez

mais à faire travailler plus longtemps les salariés. Nous vous demandons, monsieur le Premier ministre, de renoncer à ce projet dogmatique, suscitant des inquiétudes parmi nos compatriotes déjà meurtris par la crise que nous traversons. Votre label, c'est l'État et les territoires. Bien Mais jamais hier je n'ai entendu évoquer les raisons profondes de la détresse de nombre de nos communes, départements et régions : la disparition, l'effondrement du service public et l'étranglement financier. Vous évoquez même le retour du commissariat au plan. au plan. Il y a du Cervantès dans cette conviction ! Comment planifier alors que tout a été cédé aux actionnaires ? Monsieur le Premier ministre, pour planifier la reconstruction de notre économie et de notre industrie, pour mettre l'écologie

M. Macron a parlé du fret, des trains de nuit, des petites lignes ferroviaires, qu'il voulait pourtant achever avec ses bus éponymes voilà cinq ans.

solidaire et du retour à une souveraineté nationale industrielle, qui permette à notre peuple de retrouver la certitude d'un avenir. Oui, les collectivités locales, qui sont au coeur de l'organisation des différents territoires de notre pays, ont un rôle décisif à jouer.

ou presque ! Le cap est maintenu quand on entend M. Macron accepter, justifier la baisse des salaires contre la préservation de l'emploi. Du bout des lèvres, il appelle les entreprises à modérer le versement des dividendes. Mettre sur le même plan ces deux éléments dans une forme de donnant-donnant est inacceptable ! D'un côté, on réduit le revenu des salariés, souvent modestes, qui devront sacrifier des éléments essentiels de leur vie ; de l'autre, on suggère à des fortunes de limiter une part marginale de leurs revenus. Monsieur le Premier ministre, nous divergeons au moins sur deux points essentiels : il n'y aura pas de reconstruction sans répartition des richesses et sans un nouveau partage du travail. L'appellation de « Président des riches

que 800 000 à 1 million de chômeurs supplémentaires sont attendus d'ici à la fin de l'année, qu'il faut « travailler davantage », qu'il faut user et abuser des heures supplémentaires, qu'il faut rallonger l'âge de départ à la retraite ? La crise, mais aussi

de la retraite à 60 ans et de la semaine de 32 heures. C'est beaucoup ! Nous vous demandons dès aujourd'hui d'agir avec fermeté contre les entreprises qui licencient, alors qu'elles touchent des aides massives ou qu'elles réalisent des profits boursiers. Allez-vous sanctionner celles qui ont bénéficié du dispositif de chômage partiel, tout en continuant à produire ? Bien évidemment, nous approuvons l'idée de ne pas laisser sur la touche les 800 000 jeunes arrivant sur le marché de l'emploi en septembre prochain. Mais pourquoi

Monsieur le Premier ministre, pendant la guerre du Vietnam, le monde entier s'était moqué d'un commandant américain, accusé d'avoir rasé un village, qui avait eu cette explication bizarre : « Lorsque nous sommes arrivés, l'ennemi était déjà là. Pour sauver le village, nous avons dû le détruire. » Aujourd'hui, pour sauver le monde de la pandémie, il a fallu sacrifier l'économie. Voilà la situation redoutable dans laquelle vous entamez votre mandat. Autant dire que l'on vous a confié un job à 10 000 aspirines, monsieur le Premier ministre il faut toujours regarder le bon côté des choses, surtout lorsqu'il n'y en a pas ... Le temps dont je dispose étant inversement proportionnel à l'ampleur du sujet, je me bornerai à trois réflexions. Ma première remarque concerne le mythe de l'État père Noël. La France sortira essorée de la crise. Les démagogues vont se déchaîner, à commencer par les marchands d'illusion de la dépense publique illimitée, mouvement alimenté par l'improbable quatuor Soros, Minc, Pigasse, Mélenchon, ont décidé de promouvoir en commun l'idée qu'il était devenu ringard de rembourser ses dettes. Les rois d'autrefois avaient déjà trouvé une solution, qui consistait à trancher la tête de leurs créanciers. C'est vrai ! Le monde est devenu plus doux. Aujourd'hui, on nous propose seulement de les ruiner Les économistes s'affrontent désormais là-dessus sur Twitter et BFM, comme les médecins sur la chloroquine. Le principal intérêt de ces débats est de redonner des lettres de noblesse aux astrologues. ce qui est grave, c'est que cette croyance va faire déployer toutes les banderoles à la rentrée, puisqu'elle implique qu'il n'y a plus de limite au financement à crédit et à l'infini de toutes les politiques publiques. Elle renforce l'idée bien française que l'argent public est comme l'eau bénite et que chacun peut se servir. Bien sûr, pour l'heure, il n'y a pas d'autre solution que le keynésianisme sous stéroïdes adopté par le monde entier et qui nous a tellement manqué, en 2009, quand une certaine Banque centrale européenne agissait plus comme un club sadomasochiste que comme la bouée de sauvetage qui nous aurait remis à flot. à une telle solution. Mais gardons-nous de confondre plan de relance et financement de déficits incontrôlés. Sans cela, vu la dette que nous laisserons à nos enfants, nous ne devrons plus être surpris que les bébés crient à la naissance. Je dis cela, car, alors que l'on ne parle à juste titre que de l'emploi, l'on a parfois l'impression que certains de nos concitoyens éprouvent quelque peine à envisager la reprise du travail. La France possède tout de même le seul syndicat au monde ayant déposé un préavis de grève le jour du déconfinement et traîné au tribunal les entreprises qui redémarraient à grand-peine. Le Président de la République avait déclaré en avril dernier : « Il n'y a pas d'argent magique ». Puissiez-vous, monsieur le Premier ministre, tenir ce cap et expliquer sans relâche que la clé de la reprise est le travail, pas l'argent tombé du ciel. la suivante : depuis les élections municipales, nous sommes tous « écolos » ! Le bonheur est dans le pré ! C'est une excellente nouvelle. Mais quelle écologie ?

constituent un catalogue de contraintes qui sont le fonds de commerce des ONG décroissantes. La décroissance est l'opium des bobos, comme nous l'ont prouvé récemment avec éclat, en une du, dans dans une proclamation aussi subversive que du fromage à tartiner, une brochette de stars « kérosène » au bilan carbone le plus élevé de la planète. C'est risible, mais ce n'est pas drôle Ce qui est ennuyeux, c'est que la convention s'est gardée de répondre aux questions essentielles. Comment parvenir à une énergie décarbonée dans l'hypothèse où l'on décide de se passer du nucléaire ? Comment faire cesser l'hypocrisie de l'importation de millions de tonnes d'OGM, tout en interdisant les OGM à nos agriculteurs ? Comment faire payer les émissions de carbone chez nous et à nos frontières ? quelles sont les pistes pour la seule solution réaliste au défi climatique : la croissance verte, l'innovation, les nouvelles énergies, les start-up, la recherche et développement, le capital-risque, la formation La France a sabordé son industrie avec une méthode simple : tout ce qui bouge, on le taxe ; tout ce qui bouge encore, on le réglemente ; tout ce qui ne bouge plus, on le subventionne. L'Europe a raté la grande révolution des quarante dernières années, à savoir le numérique. La prochaine révolution est celle des industries de la transition écologique, que notre absence de pétrole devrait nous faire aborder avec plus d'atouts que nos concurrents, freinés par les lobbies de l'or noir. L'avenir est là, et pas dans l'écologie du « gentil avec les arbres, méchant avec les hommes » qui ne fait croître que les ronds-points. ministre -concerne les missions régaliennes. La situation est critique. Alors que de nombreuses catégories de Français, à commencer par les soignants et les premiers de corvée, ont été admirables, les droits de retrait dans l'administration ont atteint des sommets. La justice a quasiment suspendu son activité pendant trois mois, les greffiers n'ayant pas les moyens de télétravailler. Mais le dossier le plus alarmant est celui de la police. Sa crise touche aujourd'hui sa légitimité, ses doctrines d'intervention, son organisation et ses fonctionnaires. Pas de chance pour nos policiers : après le chewing-gum, le McDo, les westerns et le rock'n'roll, on importe aujourd'hui d'Amérique les névroses sur la race, qui n'ont rien à faire sur nos terres universalistes, et le pauvre policier de banlieue est désormais traité de porc, comme celui de Chicago. Il est temps que les politiques, les journalistes, les intellectuels, particulièrement ceux du « camp du bien terrorisés depuis toujours par la panique de ne pas être du côté des victimes, prennent conscience que le racisme n'est pas le fait de ceux que l'on accuse aujourd'hui, mais des faux antiracistes que sont les racialistes, les indigénistes et les décoloniaux. Écoutons la leçon de lucidité d'Abnousse Shalmani : « Une image m'a glacée lors de la manifestation pour Adama Traoré : un policier noir se fait harceler par la foule qui lui crie : " Vendu ! T'as pas honte ? " Reprocher à un homme noir d'être un policier équivaut exactement à interdire à un homme noir l'accès à la députation, à un bar ou à un mariage mixte sous prétexte de sa couleur. [ ...] Ce qui résonne dans ce discours, c'est la prison de la victimisation et l'essentialisation. » Nous attendons de votre gouvernement qu'il trouve les mots pour s'opposer à cette tragi-comédie burlesque. Autant que de moyens, les policiers ont aujourd'hui besoin de respect et de considération. considération. À ceux qui ont décidé de discréditer la police pour mieux discréditer l'État, il faut répondre que ceux qui menacent les Français, ce sont les terroristes, les criminels, les dealers et les bandes armées de kalachnikov dans les rues, mais pas la police

Si nous parvenons à convaincre nos partenaires, alors la crise du coronavirus aura pour conséquence un grand pas en avant de l'Europe. C'est pour payer l'énorme dette de la guerre contre les Anglais que les Américains ont, pour la première fois, rassemblé leurs États et lancé la marche vers les États-Unis d'Amérique pour l'Europe, ce premier pas en vue de l'harmonisation financière, budgétaire et fiscale est essentiel. Nietzsche disait : « l'Europe ne se fera qu'au bord du tombeau. Il prédisait alors les guerres à venir et la sagesse de ceux qui, après 1945, ont jeté les bases de l'Union européenne. Sa prophétie vaut aussi pour notre temps

après deux déclarations de politique générale, deux discours devant le Congrès de Versailles et une lettre aux Français qui marquaient les orientations du mandat, il vous appartient, monsieur le Premier ministre, de fixer les nouvelles priorités de l'action gouvernementale. Vous me permettrez d'en profiter pour rendre hommage à votre prédécesseur, M. Édouard Philippe, qui a dû surmonter des épreuves importantes. Il a été à la hauteur de sa tâche et, au nom de mon groupe, je voulais lui adresser des salutations respectueuses et républicaines. La période La période qui s'ouvre ne s'annonce pas des plus sereines ; il va nous falloir mettre les bouchées doubles. De la même manière qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, une pandémie ne fait pas le ménage. Depuis le déconfinement, on ne parle plus que du monde d'après, comme si la crise sanitaire avait balayé tout ce qui nous préoccupait encore il y a quelques mois. Sous le tapis Sous le tapis les gilets jaunes et leurs problèmes, les difficultés en matière de laïcité, de sécurité, d'immigration, la communautarisation de notre société sous le voile de la covid la violence, l'incivisme, la radicalité, tout ce qui sape le lien social depuis des décennies. Tôt ou tard- et plutôt tôt que tard ! -, tous ces sujets vont refaire surface ; évacués par la grande porte de la crise sanitaire, ils reviennent déjà par la petite fenêtre de l'actualité

d'abord, une crise sanitaire persistante, comme nous le rappellent nos compatriotes qui vivent à l'étranger, parce que la maladie est toujours là. La pandémie peut se raviver ici ; il faut donc rester prêt à réagir avec l'expérience que nous avons acquise. avons acquise. S'y ajoute une crise économique et sociale terrible dont les jeunes vont être les premières victimes : ils héritent de la dette sociale, de la dette environnementale et maintenant de la dette issue de la

premier axe est la relance. Ouvrir les vannes de la dépense serait inutile, puisque les ménages ont épargné, semble-t-il, entre 60 et 80 milliards d'euros durant le confinement. Dans les circonstances actuelles, relancer la demande, c'est restaurer la confiance : les gens ne consomment pas parce qu'ils ont encore peur

également le chômage, avec raison, malheureusement, puisque tous les analystes prévoient entre 800 000 et un million de chômeurs supplémentaires d'ici à la fin de l'année. C'est considérable. Restaurer la confiance, c'est donc maintenir les salariés dans l'entreprise,

trois conditions : il faut que le dispositif soit discuté et adapté par les partenaires sociaux, branche par branche, que les abus et les fraudes soient poursuivis et punis et que l'effort consenti aujourd'hui soit récompensé par plus de participation et d'intéressement pour les salariés.

Plus fondamentalement encore, rétablir la confiance impose de convaincre que l'on peut vite renouer avec la croissance. Pour ce faire, nous avons besoin d'une vision stratégique capable d'identifier les secteurs dans lesquels la France peut demeurer ou devenir leader.

Il ne faudra pas oublier le tourisme, premier secteur d'activité de notre économie, dont certaines modalités devront être repensées. C'est dans le domaine de la transition environnementale que l'on a le plus besoin d'une vision stratégique. Pour l'heure, nous ne la discernons pas

Plus fondamentalement, quelle est notre voie énergétique ? Vous n'en avez pas dit un mot. La fermeture de Fessenheim comme le maintien d'une baisse du nucléaire dans le mix énergétique entretiennent le doute. Les acteurs sérieux de l'environnement savent qu'il ne peut y avoir de transition énergétique sans le nucléaire. Nous sommes leaders dans ce domaine, mais, plutôt que de vouloir le rester, nous allons amorcer un repli. C'est difficilement compréhensible, à moins que l'on nous démontre, chiffres à l'appui, que la France pourra atteindre la neutralité carbone en 2050 tout en se dégageant de l'atome, grâce à l'hydrogène. Nous en serions heureux, mais encore faudrait-il pour cela que nous soyons capables de développer parallèlement nos énergies renouvelables dans les proportions requises,

Enfin, il n'y aura pas de relance sans solidarité, en premier lieu envers les jeunes, nous en sommes d'accord, monsieur le Premier ministre, mais aussi à propos des retraites. Or, après vous avoir écouté, je continue de m'interroger : la réforme systémique par point aura-t-elle lieu ?

Chiche ! L'attente sera forte en faveur d'un État capable de se réformer, svelte, agile et réactif. Nous nous réjouissons aussi d'apprendre que les collectivités vont être associées étroitement au plan de relance. Nous applaudissons, enfin, quand vous affirmez vouloir consacrer la différenciation, différenciation, nouvelle étape indispensable de la décentralisation. Les collectivités territoriales doivent pouvoir adapter les normes en fonction de leurs particularités et des priorités locales. monsieur le Premier ministre, « réarmer les territoires », pour reprendre vos mots, impose aussi de leur redonner de l'autonomie fiscale. Tous les volets du plan de relance doivent se tenir. Pour relancer l'économie, le Président de la République a annoncé une baisse des impôts de production. Dès lors qu'il s'agit de

cette direction, c'est-à-dire vers plus d'Europe et vers une Europe plus forte et plus unie. L'autre acteur à ne pas mettre de côté est le Parlement. Nous nous réjouissons que le Président de la République compte de nouveau sur les corps intermédiaires, puisqu'il en appelle largement aux partenaires sociaux, mais le seul corps intermédiaire oublié est, paradoxalement, le plus légitime : le Parlement. Depuis le début de la législature, nous avons l'impression d'un évitement permanent des assemblées, singulièrement du Sénat. On écoute des citoyens tirés au sort, mais on ne prête pas davantage attention aux propos de ceux qui ont été élus par les citoyens ou par leurs concitoyens eux-mêmes élus.

En effet, vous tendez la main et vous souhaitez travailler avec les élus, en partant du local. Je vois plus de régalien, de keynésien, de républicain ; on oublie la « start-up nation ». J'ai envie de vous dire : « Bienvenue en France » ! Puissent le travail du Parlement et celui du Gouvernement se conjuguer aussi souvent que possible dans l'intérêt de notre pays. Avec mon groupe, nous y sommes prêts.

de la France et que, dans la République, il n'existe qu'un seul souverain : le peuple français. C'est lui, et lui seul, que vous devez servir dans le cadre de nos institutions républicaines bicamérales,

La France dirigée par une assemblée unique ; c'est-à-dire l'océan gouverné par l'ouragan. » Ce sont nos institutions et, si vous êtes attaché à votre fibre gaulliste, vous vous en souviendrez.

entre le relèvement, qui est possible, et l'engourdissement, c'est-à-dire dire le décrochage et le déclin. Les décisions que vous serez amené à prendre dans les prochaines semaines ou les prochains mois détermineront l'avenir de notre pays, pas seulement pour ce quinquennat, mais aussi, sans doute, pour les

l'un des plus mauvais résultats dans le monde développé en matière de violence de la récession. Il faudra agir vite sur deux urgences simultanément. L'urgence sociale,

ne vous enfermez pas dans les recettes du passé, car vous ne bâtirez pas l'avenir avec de vieilles solutions, telles que des contrats aidés. Pour des jeunes qui sont souvent sans qualification, qui ont connu un échec scolaire, préférez des contrats d'apprentissage de nouvelle

qui paiera nos dettes et qui protégera les Français du déclassement et de l'appauvrissement, aussi bien collectifs qu'individuels. Pour aller chercher le potentiel de croissance, il faut toutefois agir puissamment sur deux facteurs

Je ne connais pas, ni dans nos expériences individuelles ni dans les expériences historiques collectives, de grande épreuve surmontée dans la facilité. Oui, il faudra du courage ! Il faut dire la vérité aux Français et tourner le dos à tous les mensonges qu'on leur a fait depuis des années.

est celui qui s'est le plus tertiarisé. Nous avons remplacé des salaires de 48 000 ou 50 000 euros par des salaires plus modestes dans le tertiaire.

Qui peut croire que, demain, nos créanciers n'exigeront pas le remboursement de leurs créances ? Qui peut croire

parce que tous les piliers de nos institutions, les uns après les autres, ont été ébranlés. La République est défiée à Dijon quand les différends entre bandes s'y règlent non pas au commissariat ou à la préfecture, mais dans une mosquée

! Oui, la justification de la décentralisation, c'est d'abord de recoudre le fil de la confiance dans la proximité. Avec la loi NOTRe et d'autres textes, nous avons, au

à Bayonne, d'un chauffeur de bus ! À Aiguillon ou à Bayonne, pourtant, c'est la loi de la violence ordinaire qui a prévalu. La France est désormais le pays d'Europe

de politique pénale ? Ce sont des questions concrètes auxquelles vous devrez répondre, parce que l'État a été fragilisé. Le tissu de la nation française

Si, pour être aimable, la France doit d'abord se reconnaître coupable, comment nous, Français, qui n'aurions alors de notre histoire qu'une vision lacrymale et pénitentielle, pourrions-nous nous projeter dans l'avenir pour surmonter l'épreuve ? Si l'on dit que la France est un contre-modèle,

pour dire la conviction qui m'habite : vous ne pourrez pas répondre à la dépression économique et sociale sans répondre à la dépression civique, c'est-à-dire à la défiance- cette défiance qui est fille de l'impuissance,

avec sa destinée- un peuple libre, uni face à l'épreuve, uni dans un idéal français, cet idéal qui nous rassemble, quelles que soient nos appartenances partisanes ou géographiques. C'est cet idéal français qui doit dessiner notre chemin, qui doit être notre seule perspective. Si vous empruntez ce chemin, nous serons à vos côtés ; si vous vous en détournez, nous combattrons votre politique. Vive la République et vive la France

la responsabilité qui est la vôtre, monsieur Castex, est lourde. En prenant les rênes du Gouvernement, vous avez le devoir de conduire la politique de notre pays. Cette tâche est écrasante, nous le savons, et elle revêt aujourd'hui un caractère particulier, que l'on pourrait qualifier d'historique. Historique comme la crise que nous traversons. Dans une telle période, votre rôle est de veiller à ce que les Français soient protégés, face à un virus mortel pour certains organismes, organismes, face aux conséquences d'une maladie qui mine nos habitudes, nos manières de vivre, de travailler, face à l'effondrement économique et social, qui a été abordé à plusieurs reprises dans les discours précédents, alors que les signes avant-coureurs d'une seconde vague se multiplient. Le Président de la République, qui vous a précédé dans les annonces et les déclarations, a voulu tracer un nouveau chemin et a évoqué « les jours heureux ». Aussi, c'est une déception, monsieur le Premier ministre, quand nous découvrons vos déclarations, tant à l'Assemblée nationale que, aujourd'hui au Sénat. Un élément manque, mes chers collègues : c'est l'urgence. Le groupe socialiste et républicain vous demande d'agir depuis de longs mois. Un plan de relance d'ampleur devrait être lancé ; malheureusement, à chacune de nos demandes, c'est la même rengaine : « Vous allez voir ce que vous allez voir dans le prochain

De la rapidité et des conditions mêmes de la reprise dépendront le coût économique, social et environnemental, mais aussi politique de la crise. Chaque jour perdu accroît la facture, accroît la fracture. Votre majorité en a été la première victime lors des élections municipales du 15 mars et du 28 juin

Elles ne dessinent en rien un futur rassurant pour les Français, qui subissent de plein fouet les plans sociaux et la baisse du pouvoir d'achat. Je regrette d'ailleurs que, dans vos annonces, le pouvoir d'achat soit quasiment absent, exception faite pour les personnels soignants. Après deux mois de confinement et une crise économique et sociale d'une ampleur historique, nous sommes placés face à un triple défi : soutenir le pouvoir d'achat amputé par la crise de ceux qui ont les revenus les plus modestes ; réorienter vers la consommation et l'investissement l'épargne que les ménages ont constituée pendant la période de confinement- 55 milliards d'euros accompagner les secteurs dont l'activité a été la plus affectée- je pense à l'hôtellerie, à la restauration, aux loisirs ou à la culture, monsieur le Premier ministre, un secteur qui, manifestement, vous intéresse peu, d'après vos différents discours. Pour cela, nous avons proposé un chèque « rebond solidaire » pour les ménages, mais vous ne vous saisissez pas de cette proposition. Vous préférez ne pas revenir sur la baisse des aides personnalisées au logement, les APL, alors qu'il est urgent de réaffirmer leur rôle fondamental de redistribution, de cohésion sociale et d'amortissement de la crise. Nous le savons, dans les crises, ce sont toujours les plus fragiles qui paient l'addition finale. Alors que 700 000 jeunes vont entrer sur le marché de l'emploi, vous avez axé vos annonces sur la facilitation de l'embauche des jeunes par les entreprises. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous redécouvrez manifestement l'intérêt des emplois aidés. pourquoi les avoir supprimés, ou quasiment, à partir de 2017 ? Sans chômage, sans RSA, que ce soit dans les campagnes ou dans les quartiers, les jeunes sont les plus éloignés de l'emploi et cette crise les repousse encore plus loin dans les marges de notre société. Vous annoncez, monsieur le Premier ministre, 100 000 services civiques. J'ai été ministre de la jeunesse, et je peux vous dire qu'on ne crée pas en claquant des doigts 100 000 services civiques ; ils doivent correspondre à des missions utiles pour la société. Permettez-moi de vous le dire simplement. La pauvreté n'est jamais un choix il faut la combattre. Vous avez appelé à ce que vous soient transmises des propositions. Chiche ! Nous avons une proposition : le revenu de base. Dix-neuf départements de gauche ont dit depuis deux ans leur disponibilité pour l'expérimenter : donnez-leur les moyens de le faire Dans 1 500 quartiers de la politique de la ville où ce revenu de base serait bien utile, les populations sont confrontées à une perte, voire à un effondrement de leurs ressources. L'aide alimentaire y est devenue incontournable. nationale pour la rénovation urbaine. Seraient-ils en panne ? Cette mesure est nécessaire, mais la rénovation urbaine ne doit pas être isolée d'une politique globale : il faut donner les moyens au secteur associatif, aux travailleurs sociaux et aux médiateurs de revenir activement sur le terrain et mettre en oeuvre un plan de 30 000 emplois aidés en ciblant les étudiants et les jeunes dans les quartiers. La remise en cause drastique et brutale de ces contrats a été une erreur, monsieur le Premier ministre. Reconnaissez-le. Ils constituent un levier de soutien fort et rapide, facilement mobilisable. Autre absent de taille : vous avez peu parlé de l'Europe, finalement, tandis que se jouent aujourd'hui les négociations sur le plan de relance européen et le cadre financier pluriannuel. Alors que la France sera l'un des pays les plus touchés par la chute attendue de son PIB, pourquoi attendez-vous septembre pourquoi attendez-vous septembre pour mettre en place un plan de relance ? Une partie de nos partenaires agissent vite, parfois même, comme en Allemagne, en tournant le dos aux politiques anciennes. En France, finalement, pour Emmanuel Macron, la seule rupture politique a été de changer de Premier ministre. Le Président de la République est passé de l'art du « en même temps » à l'art du contretemps. La seule rupture que nous observons avec ce gouvernement concerne peut-être la grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes, qui a dû s'effacer devant les équilibres politiques nécessaires pour former le Gouvernement Nous aurons l'occasion de vous interroger tout à l'heure sur ce sujet dans le cadre des questions d'actualité. Plutôt que de la rupture, je vois de l'immobilisme, un immobilisme coupable quand il concerne des réformes qui ont fragmenté notre pays et fragilisé les plus faibles. Aujourd'hui, votre rôle, monsieur le Premier ministre, est de rassembler les Français, de les protéger, de les accompagner face à cette crise, mais certainement pas de relancer la réforme des retraites, qui a déjà laissé tant de traces. Des centaines de milliers de Français sont descendues dans la rue pour lutter contre les mesures contenues dans ce texte. Le chiffon rouge de l'âge pivot sera peut-être retiré, mais la cicatrice de l'article 49, alinéa 3 sera toujours présente. Ce projet a également suscité une forte opposition des syndicats, ouvriers comme patronaux. Permettez-moi de m'étonner, monsieur le Premier ministre, alors que vous prêchez « le dialogue, l'écoute, la recherche du compromis », que vous que vous annonciez la reprise de cette réforme, dans une logique, permettez-moi de le dire, d'obstination décalée eu égard à la situation. En faisant cela, vous remobiliserez les forces vives de notre pays contre un projet inique que vous auriez dû finalement abandonner, afin de ne pas pas pénaliser une nouvelle fois l'économie face à une forme de cataclysme social qui s'annonce. Il en est de même de l'assurance chômage : votre réforme, celle qui est venue et celle qui vient, est très dure pour les Français les plus modestes. Le contexte économique et social dans lequel la pandémie nous a plongés la rend aujourd'hui particulièrement dangereuse. Je vous demande, monsieur le Premier ministre, au nom de mon groupe, non pas de l'amender, de la faire évoluer, mais de l'abroger purement et simplement. L'environnement doit être aussi un axe fort du plan de relance. Vous avez raison : la rénovation énergétique des logements est indispensable. Le bâtiment représente 43 % de la consommation d'énergie finale en France et compte pour près du quart des émissions de gaz à effet de serre. C'est un gisement majeur de bénéfices environnementaux, économiques et sociaux. Malheureusement, le dispositif que vous proposez nécessite une avance que de nombreux propriétaires ne pourront pas faire. Il faut démocratiser la rénovation thermique, en instaurant une « prime climat » qui permettra un préfinancement public et qui s'adaptera au niveau de revenus des propriétaires. Cette crise est également l'occasion de repenser notre modèle et d'aller vers plus d'indépendance. Nous avons pu constater que la France n'était pas en capacité de répondre, à titre individuel, à l'urgence sanitaire. Manque de respirateurs, manque d'équipements de protection, manque de certains médicaments : cette crise a été un révélateur, ce dont, je crois, vous avez pris conscience. Comme nous tous ici dans cette Haute Assemblée, vous partagez ces constats, mais de Luxfer, de Famar ? Les déclarations d'intention, c'est bien, monsieur le Premier ministre, mais cela ne suffit pas : il nous faut des actes, et je crains que nous ne les attendions encore longtemps. Depuis trois ans, votre majorité mène une politique plus bénéfique aux très riches et aux multinationales qu'elle n'est favorable aux précaires et aux PME françaises. Suppression de l'ISF, mise en place de la, suppression de l', baisse de l'impôt sur les sociétés pour les grandes multinationales, suppression de la taxe d'habitation pour les 20 % de contribuables les plus aisés : la liste est longue. J'ai bien entendu le Président de la République,

même si nous comprenons que, finalement, la taxe d'habitation pourrait être un outil utile pour l'ensemble des Français quand il s'agit finalement de financer les services publics locaux. En tout cas, demander aux entreprises de baisser les dividendes sans Demander des dons en faveur de l'hôpital public sans créer un nouvel impôt sur le capital, comme nous vous l'avons proposé, ne suffira pas, et cela ne trompe personne. D'ailleurs, la vraie question, monsieur le Premier ministre, qui va payer et dans quelles conditions allez-vous assurer la redistribution dans notre pays pour faire face à la crise et aux dépenses que vous avez décidé d'engager ? Enfin, cette solidarité que nous appelons de nos voeux doit être territoriale. Il faut d'urgence porter secours à nos territoires les plus fragiles. Je pense à la Guyane, où vous étiez il y a quelques jours. Ce sont ces territoires,

qui sera, je l'espère, le vôtre en matière de décentralisation. Il est vrai que vous parlez beaucoup de territoires. Je crois que vous avez cité ce mot une cinquantaine de fois depuis hier. On peut sauter comme un cabri et prononcer ce mot. Mais tout ne viendra pas les territoires. D'ailleurs, je tiens à vous le dire, la notion de territoire pertinent, c'est un peu comme l'horizon : plus on s'en approche, plus il s'éloigne Tous les territoires ne viendront pas à notre secours. Il faut leur donner des moyens. Le groupe socialiste a fait des propositions utiles, que je tiens à vous rappeler. La priorité doit être de clarifier la répartition des compétences au sein de la République. L'État doit enfin mener à bien la réforme de sa propre organisation déconcentrée et permettre l'autonomie des collectivités. Derrière le mot « autonomie », je place l'expression fiscale, monsieur le Premier ministre. L'autonomie fiscale n'est pas un gros mot, et je la préfère à la notion d'autonomie financière, soutenue par le Président de la République, qui aboutit finalement au contrat de Cahors, un contrat scélérat au regard de la décentralisation- je vous le dis ici haut et fort, à cette tribune. L'autonomie fiscale, c'est finalement permettre aux collectivités de décider librement ce de décider librement ce qu'elles ont envie de faire pour leurs concitoyens, sous le contrôle démocratique qui intervient tous les six ans pour les communes, les départements et les régions. La liberté des collectivités territoriales, c'est l'article 72 de la Constitution, et les conditions y sont clairement identifiées. Pour passer le cap d'une rentrée économique et sociale qui sera difficile, monsieur le Premier ministre, il faut urgemment prolonger le plan de soutien aux collectivités par un « plan de rebond territorial ». Cette relance que j'appelle de mes voeux passera par les élus locaux. Pour cela, il convient de ne pas avoir de tabous, de les doter de plus de leviers d'action : plus de subsidiarité, plus d'expérimentations locales, plus de différenciation, plus de pouvoir réglementaire, plus d'interterritorialité, pour leur permettre d'exister face à un État qui, aujourd'hui, a besoin de partenaires. Vous l'avez compris, le groupe le groupe socialiste et républicain ne peut pas trouver son compte dans votre déclaration, dans vos déclarations de politique générale. D'ailleurs, je crois que vous avez eu une bonne idée en ne demandant pas la confiance au Sénat. Vous appelez à la concorde nationale, mais celle-ci ne se construit pas dans l'amnésie générale, dans l'anesthésie générale que portent finalement vos déclarations et encore moins dans l'amnistie générale pour les trois années qui ont précédé votre propre prise de responsabilités à Matignon. Monsieur le Premier ministre, nous serons donc une opposition vigilante, exigeante, constructive et j'espère que, de temps en temps, vous saurez écouter votre opposition pour faire progresser votre politique nationale, au service des Français et de notre pays.

peu importent les qualificatifs, votre nomination intervient à un moment particulier, celui de la pire crise sanitaire qui nous a frappés en un siècle. Elle inaugure aussi un nouveau cycle de la vie politique de notre pays, dont l'horizon aura pour terme l'élection présidentielle de 2022. Nouvelle illustration, s'il le fallait encore, que la V République telle que nous la vivons doit être profondément repensée pour en casser la verticalité, pour réhabiliter les corps intermédiaires ou donner plus de souffle à la démocratie locale. Or l'accélération des cycles politiques imputable à l'instauration du quinquennat, renforcée par le prêt à penser en 280 signes et le diktat médiatique, fait qu'il est de plus en plus difficile de bâtir et de tenir une vision de long terme pour notre pays. Il faut bien le constater : notre société est psychologiquement épuisée après une succession de crises majeures. La peur de l'avenir paralyse les initiatives et tétanise notre jeunesse. Le sentiment de déclin est prégnant. Notre économie connaît ses pires moments depuis des décennies. Les fractures identitaires gangrènent de plus en plus de zones, quand d'autres territoires excentrés se sentent oubliés. Votre feuille de route est un immense défi, à l'image de l'ambition que nous devons avoir pour la France : reconstruire une confiance durable entre les citoyens et leurs gouvernants pour relever notre pays. Nous n'avons pas le droit de céder au défaitisme, car la République, notre bien commun, doit être défendue chaque jour. Fort de la liberté d'esprit, de ton et de vote qu'il a toujours cultivée, mon groupe, le RDSE, entend soutenir tout ce qui contribuera à ce relèvement, par-delà les attaches partisanes, sans subir la pression de la rue ou des réseaux sociaux. Au nom du seul intérêt général. Redonner confiance à nos concitoyens, c'est d'abord agir par des mesures simples et concrètes pour leur quotidien. Ce que mon groupe attend, c'est que la promesse républicaine d'égalité soit une réalité. La crise sanitaire a montré que notre modèle social fonctionnait, n'en déplaise à ceux qui n'en regardent que le coût. Il faut maintenant aller plus loin sur le plan social pour « bâtir les fondations de la France de demain », comme vous l'avez dit. Face à l'explosion de la précarité et du chômage, votre gouvernement se doit d'agir avec efficacité, afin de mieux accompagner les plus vulnérables et d'offrir, à tous, les mêmes chances de réussite. Tous ceux que la crise a frappés de plein fouet, pour qui ce virage social est indispensable. La crise des « gilets jaunes » l'a bien souligné : nos concitoyens attendent avant tout une véritable justice sociale, notion que l'on ne saurait réduire à de l'assistanat. Mon groupe y attache une importance fondamentale. Il est temps, par exemple, que le plan Pauvreté tant de fois annoncé se concrétise ! Vous avez également déclaré vouloir promouvoir l'approche par les territoires, et je sais que cet hémicycle vous a écouté d'une oreille très attentive. Monsieur le Premier ministre, mon groupe a envie de vous prendre au mot, quand on sait que nos collectivités n'en peuvent plus de cette instabilité normative désespérante. Et bien sûr sans les financements qui permettraient d'y faire face Pourtant, la crise sanitaire a révélé de formidables initiatives des élus locaux, avec, très souvent, des préfets pleinement investis pour les soutenir. Allons plus loin pour une organisation encore plus vertueuse, avec une déconcentration d'abord soucieuse de l'efficacité et des spécificités locales- plutôt que d'en référer en permanence à Paris -, une décentralisation qui ferait confiance aux élus et qui leur permettrait de mettre en oeuvre une véritable différenciation dans le respect des libertés locales et de l'unité de la République. La réalité est tout autre. Nous le constatons quand nous croisons dans nos territoires beaucoup de souffrance et d'incompréhension, du fait de l'abandon de l'État : dans les zones rurales enclavées qui subissent les fermetures de services publics, dans les zones urbaines victimes de retards économiques et sociaux accumulés, dans les zones périurbaines, indispensables pourvoyeuses de main-d'oeuvre, mais toisées par des métropoles devenues inaccessibles sur tous les plans. Monsieur le Premier ministre, mon groupe est totalement investi pour défendre la dignité de nos compatriotes. Il ne saurait exister de citoyens de second rang du fait de leur lieu de résidence. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons proposé la création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, avec comme ambition de créer un outil au service de toutes les collectivités. Malheureusement, l'ANCT n'a pas répondu à ces objectifs, se transformant en une machine administrative obèse et édulcorée comme notre technocratie en a le secret. L'égale dignité de nos concitoyens, c'est encore assurer le désenclavement de certains territoires, pour lesquels une ligne aérienne ou une desserte ferroviaire sont indispensables sur le plan économique. Nous comptons sur vous pour soutenir les collectivités et garantir le respect des obligations de service public des opérateurs. Je pense en particulier à l'aérien. Très bien ! Vous avez aussi annoncé vouloir réhabiliter les trains de nuit, les petites lignes et le fret ferroviaire. Nous ne pouvons qu'approuver, à la condition toutefois qu'il ne s'agisse pas de promesses non suivies d'actes. Il y va de l'attractivité, voire de la survie de nombreux territoires Cela vaut tout autant pour le numérique, alors que la crise sanitaire a révélé de profondes inégalités en la matière. Mon groupe travaille en particulier pour que l'accès au très haut débit soit une réalité partout, mais aussi pour que la lutte contre l'illectronisme devienne une grande cause nationale, à la suite des travaux de la mission d'information dont nous sommes à l'origine. Cela vaut encore en matière d'écologie, avec les défis immenses qui nous attendent et pour lesquels nos concitoyens sont prêts à changer leurs habitudes. Cela suppose toutefois de ne pas enfermer l'écologie dans une approche punitive, qui aggraverait les fractures sociales ou territoriales et servirait de prétexte à entraver le progrès technologique. Monsieur le Premier ministre, si mon groupe cultive la liberté de vote, il ne transigera jamais sur la défense de la laïcité. Vous avez raison de dire que « la République, c'est la laïcité comme valeur cardinale, comme fer de lance de la société ». Face aux velléités séparatistes, face à ceux qui veulent réécrire l'Histoire, il faut affirmer, sans jamais faiblir, que la laïcité est un facteur d'émancipation garantissant à chacun le droit de croire ou de ne pas croire. Aucune religion ou communauté ne peut revendiquer sa supériorité à la loi commune. C'est bien pour cela que la laïcité contribue à la concorde civile et à l'unité de la Nation, car elle rend les citoyens égaux devant la loi et dans la dignité. Nous serons donc à vos côtés pour faire respecter l'ordre public face à ceux qui défient l'autorité de l'État ou revendiquent de s'extraire de la loi commune. Il est encore temps d'agir avec force La situation est grave, chacun le sait, mais nous devons nous réunir pour faire en sorte que la République demeure une et indivisible ! Monsieur le Premier ministre, vous vous êtes présenté comme un homme de dialogue et de concertation. Nous espérons que, avec votre gouvernement, vous appliquerez à la lettre cette méthode dans vos rapports avec le Parlement, en particulier Pour l'heure, et dans sa diversité et sa liberté, le groupe RDSE continuera à placer l'intérêt général de notre pays par-dessus toutes les contingences partisanes.

La parole est à M. François Patriat, pour le groupe La République En Marche. En Marche. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, dans cette dramatique crise sanitaire, vous avez, monsieur le Premier ministre, rappelé le rôle primordial qu'ont assuré celles et ceux qui, jour après jour, ont oeuvré avec courage pour sauver des vies, des milliers de vies. Face au risque réel de deuxième vague, le devoir de responsabilité que vous avez appelé de vos voeux s'impose à chacun d'entre nous. Collectivement, en tant que législateur, nous avons contribué à l'élaboration de politiques publiques efficaces. Au-delà de nos obédiences ou chapelles politiques, nous avons su être à la hauteur des enjeux. Je tiens, à cette occasion, à rendre hommage au Premier ministre Édouard Philippe, votre prédécesseur, pour le travail considérable qu'il a mené avec l'ensemble des membres de son gouvernement, avec méthode, pédagogie et détermination, sur le front de la lutte contre la propagation du virus, sur le front de la sauvegarde de l'emploi et sur le front du soutien aux plus vulnérables. Dès le début de la crise, un ambitieux plan d'urgence a été enclenché. Ainsi, 430 milliards d'euros ont été déployés, avec le recours massif au chômage partiel, les prêts garantis par l'État, la mise en place du fonds de soutien et de solidarité et une panoplie de mesures sectorielles sans lesquelles des pans entiers de notre économie auraient été réduits à néant. Je pense à l'aéronautique, à l'automobile, à l'hôtellerie, à la restauration, à la culture, et à bien d'autres encore. Je tiens également à féliciter les élus locaux qui, tout au long de la crise, ont su illustrer leur rôle d'acteurs de proximité. Chacun d'entre nous, par nos échanges et nos contacts permanents avec eux, peut en témoigner : ils n'ont jamais ménagé leurs efforts. ont invariablement su répondre à l'urgence pour repenser la vie de leur territoire au service de nos concitoyens. Oui, les collectivités territoriales sont les maillons essentiels de la reprise. Alors que les réformes ambitieuses menées par le Gouvernement pendant trois ans avaient permis au chômage d'atteindre son plus bas niveau depuis dix ans, au pouvoir d'achat de connaître sa plus forte progression et à notre pays de figurer parmi les plus attractifs nous avons su combattre ce virus avec réactivité et faire face aux difficultés. La crise a révélé nos forces, mais également nos faiblesses. Notre système de soins a tenu bon, lorsque celui de certains de nos voisins a fait défaut. Dans le même temps, la crise a révélé nos fragilités, parmi lesquelles notre trop grande dépendance aux industries étrangères, notamment dans des secteurs stratégiques. Mais l'heure n'est pas au bilan, elle est à l'action. vous avez reçu la mission d'organiser le déconfinement, avec une feuille de route précise, des étapes scrupuleusement respectées, un travail de pédagogie et un sérieux largement appréciés. Ce sérieux, nous le devons à tous les Français qui, durant de longs mois, ont accepté de restreindre leurs libertés. C'est ce sens de l'intérêt général dont ont fait montre les Français qui doit nous inspirer et guider nos choix. De par votre expérience d'élu local, vos compétences reconnues au-delà des clivages politiques, vous avez mené à bien, en lien avec les collectivités territoriales, les services de l'État et les élus locaux, une stratégie de déconfinement qui s'annonçait pourtant périlleuse. Vous avez permis une reprise progressive de nos déplacements, de nos activités, de ce vivre ensemble à la française auquel nous sommes attachés. Pour que cette reprise perdure, nous devons faire preuve à la fois de solidarité, d'inventivité et de responsabilité. La crise économique qui se profile a renforcé, chez les Français, cette peur du déclassement aux quatre coins du territoire national. Cette crise doit donc être l'occasion de réconcilier nos territoires, avec l'ambition de restaurer la confiance de nos concitoyens les uns envers les autres. La République une et indivisible ne doit pas demeurer un vain mot. Elle doit s'incarner dans les actes que nous mènerons ensemble, collectivement. Chacun d'entre nous doit prendre pleinement conscience de la gravité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Oui, mes chers collègues, nous sommes à la croisée des chemins. Soit nous agissons collégialement pour lutter efficacement contre les fragilités économiques, les situations sociales délicates, les difficultés rencontrées par nos concitoyens, soit nous sombrons dans le pessimisme mortifère, l'invective permanente, le culte de la division et de l'opposition. Sachons être dignes des exigences légitimes des Français, qui attendent de nous, élus de la Nation, un esprit de concorde, de construction commune, en faveur du seul intérêt qui compte : celui de notre pays. Pour ce faire, nous devons faire preuve d'humilité, rappeler ce qui a été réalisé depuis le début de la crise, mais également faire le point sur nos actions, sans craindre le jugement hâtif ou partiel de ceux qui pensent pouvoir faire mieux, davantage, tout le temps et dans tous les domaines.

sont confrontés aux difficultés que vous avez évoquées dans leur travail, dans leur santé, dans leurs déplacements. Ce sont ces réponses concrètes que j'ai entendues aujourd'hui. Sachez que que je ne crois pas à l'uniformité des politiques publiques, sorte de maladie qui a frappé notre pays tout au long de son histoire récente. C'est en raison d'une approche monolithique des difficultés rencontrées, comme des solutions envisagées, que nous avons été dans l'incapacité de penser un modèle d'inclusion qui puisse satisfaire l'ensemble de nos concitoyens, de Brest à Strasbourg, du Havre à Prades. À ce titre, Monsieur le Premier ministre, vous avez exprimé votre soutien au droit à la différenciation, que vous souhaiteriez voir consacré dans une loi organique. Farouche partisan de la décentralisation, je suis persuadé que nous devons entamer une nouvelle étape de celle-ci. La reprise économique et la lutte contre les inégalités sociales ne pourront être permises que si les territoires en deviennent les acteurs centraux. Vous avez fixé un cap tracé un chemin. La gestion à court terme des crises ou d'autres urgences ne peut être l'apanage d'une politique qui se veut ambitieuse. Notre politique doit s'inscrire dans le temps long : celui de la réflexion, de l'anticipation et de l'action. Comme l'a rappelé Emmanuel Macron à l'occasion de son intervention télévisée, nous devons définir une perspective, engager des réformes nécessaires à la survie de notre système dans la concertation, l'écoute et le respect du travail en commun. Identifier les secteurs d'avenir, investir dans la transition énergétique, préparer un plan pour la jeunesse : tels sont les chantiers que vous annoncez et que nous soutiendrons. Vous avez parlé des retraites, monsieur le Premier ministre. Cela fait trente que nous reculons sur ce problème ! Comme si rien n'avait été fait avant ! Au moment où nous voulons engager une réforme ambitieuse et équitable, devrait-on une fois encore reculer, parce que ce ne serait pas encore le moment ? Je crois que le Gouvernement a raison de vouloir insister et mener à bien cette réforme aujourd'hui, dans la justice sociale et dans l'efficacité. Nous nous réjouissons que les collectivités territoriales, les partenaires sociaux et les citoyens soient pleinement associés à la mise en oeuvre concrète de cette reconstruction. Oui, nous ne pourrons agir les uns sans les autres, vous l'avez dit : les élus sans les administrés, les villes sans les campagnes, les entreprises sans les salariés et réciproquement. J'en ai la certitude : la reconstruction sera le fruit d'un travail collectif ou ne sera pas. Vous avez présenté et détaillé les principaux axes du plan de relance. Vous avez évoqué

Le soutien aux secteurs en difficulté, la prise en compte des enjeux démocratiques du futur et la valorisation du dialogue social sont autant d'outils efficaces dans cette période de crise à laquelle nous sommes quotidiennement et collectivement confrontés.

Investissement et transformation seront les maîtres mots de l'action du gouvernement que vous avez l'honneur de diriger, monsieur le Premier ministre. Nous nous en réjouissons. Je retiendrai deux éléments fondateurs de votre intervention une ambition claire et une obligation de résultat concret. Ce sont notre détermination, notre énergie et notre capacité à rebâtir qui permettront à notre pays de relever les immenses défis qui se présentent à tous.

monsieur le Premier ministre.

ne me surprend pas. Ne doutez pas, mesdames, messieurs, de notre détermination très forte dans ce contexte si particulier à vouloir poursuivre et accélérer la relance de notre économie. Tel est notre premier objectif. Je n'ai d'ailleurs pas perçu

la plus riche en emplois, la plus tournée vers la transition écologique -, ni sur le contenu de nos propositions que la concertation améliorera, ni même sur la méthode que j'ai proposée, à savoir le dialogue, la proximité et le pragmatisme. J'ai entendu

vers la croissance, l'amélioration de la compétitivité de notre économie et la formation des hommes et des femmes de notre pays.

est sans doute le bien le plus précieux de notre système de protection sociale et de cohésion nationale. Absolument dans les circonstances que nous venons de traverser eut été une erreur profonde. Revendiquons ensemble cette reconnaissance juste de la Nation à l'égard de tous ces personnels.

à la gestion de la précédente crise de 2008-2010. Je l'ai vécue de l'intérieur. Elle était difficile, et l'on explique, hélas à juste titre, que celle dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui sera beaucoup plus forte. Je perçois toutefois une différence,

dans la gestion de la crise de 2008, malgré les efforts alors déjà déployés par la France. Quelque 35 milliards d'euros du plan de relance que nous vous soumettrons sont financés par l'Europe. C'est une différence majeure, à laquelle, je me permets de vous le rappeler, la France et le Président de la République ont

la perspective d'utiliser cette crise comme une opportunité. Cela vaut aussi pour l'Europe, qui doit retrouver à cette occasion de la crédibilité auprès de nos concitoyens.

conscience de la nécessité de lutter avec nous contre la crise, de se mobiliser, comme beaucoup l'ont fait dans la dimension sanitaire de cette dernière. Pour cela, il nous faut retrouver, à l'occasion de cette crise, les bases de la confiance.

de respect de la laïcité républicaine, d'écoute, de sens des responsabilités, de courage dans la conduite de réformes indispensables à notre pays.

assurés que je ne perds pas de vue l'immensité de la responsabilité qui pèse sur mes épaules. Mais c'est précisément parce qu'elle est immense